Cet article tel que rédigé repose sur la reprise d'un seul des trois éléments constitutifs de la recommandation de la mission, qui avait été conçue comme un tout. Le choix du seul forfait de réorientation, qui fait l'économie d'une réflexion plus générale sur le mode de financement des urgences, ne saurait constituer qu'une solution de " bricolage " transitoire venant complexifier encore la tuyauterie du financement des services d'urgences, sans y apporter de solution de redressement pérenne. » Je rappelle que cette proposition n° 1 envisageait la conservation d'un financement mixte incluant une part de financement à l'activité et une part forfaitaire, la modulation la modulation du montant du financement à l'activité en fonction de la gravité des pathologies et de la technicité des actes réalisés et, enfin, la création d'un forfait de réorientation visant à inciter les services à réadresser les patients ne nécessitant pas de prise en charge hospitalière vers les acteurs de ville de la prise en charge en urgence.

Comment ignorer que beaucoup de patients se rendent aux urgences, car ils n'ont pas d'autre solution médicale ? Comment ignorer les difficultés financières de nombre d'entre eux, ce qui entraîne un accroissement du nombre de renoncements aux soins ? L'accueil de chaque patient faisant partie intégrante

sur l'article. Pour appuyer les propos de ma collègue Laurence Cohen, je souhaiterais vous parler d'un bassin de vie qui rassemble 700 000 personnes à une heure de Paris. Dans le département du Pas-de-Calais, ce que nous appelons le bassin minier que nous appelons le bassin minier est en souffrance sur bien des points. En termes de santé, la situation sanitaire y est révoltante. On meurt plus à Lens qu'ailleurs. La surmortalité ou mortalité évitable y est de 76 % supérieure à la moyenne nationale. Les causes de cette de cette hécatombe sont multiples : on pourra citer les addictions pour se donner bonne conscience, mais la prévention y est très en retard, notamment en ce qui concerne les dépistages des cancers. Le peu de médecins, la saturation des hôpitaux, la situation sociale dégradée de la population sont surtout à mettre en cause. Cet article propose de réorienter les patients accueillis aux urgences vers la médecine de ville en fonction de leur pathologie. Mais si la médecine de ville était suffisante, les patients n'iraient pas s'entasser parfois plus de vingt-quatre heures aux urgences ! À Lens, l'hiver dernier, la combinaison gel plus grippe complètement saturé les urgences, les soignants étant obligés de planter des clous dans les couloirs pour suspendre les perfusions. Les personnels sont exténués. Le non-recours aux soins devient la règle. Des personnes âgées préfèrent rester chez elles plutôt que de se laisser transférer à l'hôpital et ne se soignent donc pas du tout. Les services du SMUR ont été complètement déshabillés limitant la possibilité d'intervention, à tel point que, lorsque vous êtes venue la semaine dernière, madame la ministre, vous avez insisté sur l'urgence de rouvrir la deuxième équipe du SMUR,

de grandes théories. Une maman qui se présente aux urgences le soir avec son enfant qui a mal à l'oreille et 39 de fièvre, ce n'est pas une urgence ; c'est une consultation non programmée.

On a fait l'erreur, à un moment donné, de supprimer du code de déontologie l'obligation, pour les praticiens, de s'inscrire à un tableau de garde. Chaque métier a ses contraintes- la contrainte et la grandeur, soit dit en passant, des médecins, c'est de participer de cette logique.

Les conséquences de cet article peuvent être extrêmement graves pour la santé des Français, sous couvert de vouloir réduire le temps d'attente dans les services d'urgences hospitalières. en établissant un nouveau mode de tarification aux urgences, qui pourrait s'élever de 20 à 60 euros par établissement et par réorientation de patient vers un médecin de ville pour une consultation ultérieure ou bien au sein d'un autre service hospitalier, deux risques sont encourus. Le premier est d'envoyer un mauvais signal comptable ; le second risque est médical, car si, pour certaines pathologies simples, le dispositif peut être pertinent, comment prendre la décision de réorienter certains patients et avoir la certitude que toute urgence vitale est écartée, d'autant que, lors des passages aux urgences, les antécédents et les informations de santé sont généralement parcellaires ? l'article est lui-même parcellaire, puisque se pose la question de la responsabilité de la direction des établissements de soins et des personnels soignants. Sur qui reposeront les conséquences d'une éventuelle erreur de diagnostic ou de posologie pour un traitement ou bien d'un retard de prise en charge dû à la réorientation chez un médecin de ville plusieurs jours après le passage aux urgences, qui aura peut-être fait perdre un temps précieux dans la réalisation du diagnostic En théorie, si le refus de réorientation par le patient est prévu, la pratique ne laissera guère le choix et sera source d'une prise en charge complexifiée. La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter

la conservation d'un financement mixte incluant une part de financement à l'activité et une part forfaitaire ; la modulation du montant du financement à l'activité en fonction de la gravité des pathologies, afin d'inciter les services à se concentrer sur la prise en charge des patients classés CCMU 3, 4 ou 5 ; la création d'un forfait de réorientation visant à inciter les services à réadresser les patients ne nécessitant pas de prise en charge hospitalière vers les acteurs de ville. Le dispositif qui a été présenté à l'Assemblée nationale par le rapporteur général Olivier Véran apparaît problématique à quatre titres au moins. En premier lieu, il reprend un seul des trois éléments constitutifs de la recommandation de la mission, qui avait été conçue comme un tout. Le choix du seul forfait de réorientation, qui fait l'économie d'une réflexion plus générale sur le mode de financement des urgences, ne saurait constituer qu'une solution de « bricolage » transitoire venant complexifier la tuyauterie de financement des services d'urgences sans y apporter de solution de redressement pérenne. En deuxième lieu, le dispositif pose une question d'organisation des soins. Quand bien même la réorientation du patient passerait par une consultation préalable, cette réorientation s'analyse au total comme un acte médical non accompli et pour autant rémunéré.

20 et 60 euros, selon les informations transmises par la DSS. De plus, comment le professionnel de ville sera-t-il incité à dégager son planning pour accueillir un patient venu des urgences ? du dispositif devrait reposer sur une coopération forte entre la ville et l'hôpital, dont les contours restent encore largement à construire. Pour l'ensemble de ces raisons, même si cette solution

d'urgentistes. Nous sommes passés à plus de 400 internes formés par an depuis la réforme du troisième cycle des études de médecine. La réforme holistique vise donc à travailler sur l'amont, sur les urgences elles-mêmes et sur l'aval. À cela s'ajoute la proposition d'Olivier Véran.

Ce n'est pas très incitatif d'être pertinent dans notre métier. Quand on veut changer les modes de tarification, il faut donc accepter de financer ceux qui ne font pas, parce que, pour la personne qui va renvoyer quelqu'un en disant « vous n'avez rien à faire aux urgences, on va vous trouver une maison de santé pluriprofessionnelle ouverte dans votre quartier »,

d'une entorse de cheville banale ! Quand il existe une offre de soins non programmés accessibles, il me paraît de bonne pratique de réadresser les malades. J'ai entendu que vous souhaitiez

Notre commission ne peut que souscrire aux objectifs visés : la garantie de la sécurité et de la qualité des soins dans les services hospitaliers, qui est une impérieuse nécessité. Le mécanisme prévu par cet article, à savoir la possibilité de récupérer auprès des établissements de santé les sommes indûment facturées au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d'autorisation, constitue un instrument supplémentaire pour inciter les établissements à respecter les seuils d'activité. Cependant, on comprend mal que des établissements puissent continuer de pratiquer des activités de soins sans respecter les seuils d'activité de sécurité. Pourquoi proposer une mesure financière plutôt que la fermeture de services qui n'offrent pas toutes les garanties de sécurité ? Par ailleurs, on se demande comment des procédures de contrôle pourraient être plus efficaces en matière financière si elles ne permettent pas aujourd'hui d'intervenir auprès des établissements problématiques. Il me semble donc que c'est plus sur la bonne conduite des contrôles qu'il conviendrait de se pencher. Or les modifications apportées par l'ordonnance du 3 janvier 2018 au régime de visite de conformité des ARS nous conduisent à nous interroger sur la volonté de s'assurer du strict respect de ces règles par les établissements de santé. Ces visites devaient jusqu'alors être obligatoirement réalisées dans les six mois suivant la délivrance d'une autorisation d'activité d'activité ou d'équipement ; elles sont désormais facultatives. En outre, les auditions ont fait émerger la question de l'adéquation de la définition des seuils fixés par voie réglementaire avec les conditions réelles de l'activité des établissements de santé. En effet, la définition du seuil se fait au niveau de l'établissement, mais elle ne rend pas compte en particulier de la réalité de l'activité pratiquée de manière individuelle

concerne un sujet sur lequel nous butons depuis de très nombreuses années. Il apparaît dans la littérature internationale que, pour un certain nombre de cancers, le fait d'être opéré soit par un chirurgien qui n'a pas l'activité suffisante, soit par une équipe insuffisamment formée, soit par un hôpital ne disposant pas du plateau technique adapté- cela dépend du type de cancer

Nous avions alors indiqué que ces activités ne pouvaient pas être réalisées en dehors des établissements ayant un seuil d'activité suffisant.

Mme la rapporteur.

sur les fermetures d'établissements et de services de santé. Je vous ai entendue, comme tout un chacun, madame la ministre, dire sur ministre, dire sur France Info que la réforme du système de santé ne prévoyait aucune fermeture d'un hôpital de proximité, ajoutant même qu'il y avait un mythe autour des fermetures des services d'urgences.

que la fermeture des services de l'hôpital et de la maternité est un mythe ? Pouvez-vous dire aux parents d'enfants malades de l'hôpital Raymond-Poincaré à Garches que les suppressions de lits sont un mythe ?

avant de fermer un service ou un hôpital, en engageant une concertation avec les personnels, avec les patients, en vue de trouver les solutions qui s'imposent. Or ce n'est pas le cas aujourd'hui.

Le seul engagement que je prends devant les Français, c'est de leur assurer la même qualité de soins que celle que je demande pour ma famille.

je suis défavorable à cet amendement.

3 500 accouchements pour 7 salles d'accouchement. Pour moi, c'est la chaîne.

sur les territoires français, vous creusez les inégalités en matière d'accès aux soins. Jean Lassalle vous l'a dit avec beaucoup de force- je n'ai pas son talent, et je ne chanterai pas dans l'hémicycle

est trop éloigné, ils ne peuvent pas prendre en charge les patients en première instance. Si l'on ne peut pas transférer le service des urgences dans leur périmètre d'activité, ils se trouvent dans des situations beaucoup trop difficiles en termes d'assurances et de sécurité dans l'exercice de leur profession, et on perd directement notre attractivité. On ne peut donc pas faire venir des généralistes si les urgences

Mme Troendlé ont pris la parole pour protester contre la fermeture de services de maternité en Alsace. Que je sache, la caisse d'assurance maladie d'Alsace n'est pas déficitaire, contrairement à

je tiens à rassurer les quelques-uns d'entre vous qui ont affaire à la transformation de services d'obstétrique en services de périnatalité. Un service de périnatalité,

ce projet de loi de financement de la sécurité sociale nous conduisent à penser qu'il n'y a pas lieu de changer le mode de financement de l'École des hautes études en santé publique, l'EHESP, et du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique

qui ont décidé de boycotter nos hôpitaux publics. À mon sens, cette attitude n'est pas déontologique. C'est un rapport de force qui s'est engagé. Pour l'instant, je tiens bon.

un nouveau médecin libéral ne peut s'installer en étant conventionné à l'assurance maladie que lorsqu'un médecin libéral de la même zone cesse son activité. Le principe de la liberté d'installation demeure donc, mais le conventionnement n'est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations. Il s'agit bien de traiter une problématique profonde de nos territoires, notamment ruraux. Je veux bien sûr parler de la désertification médicale ; il n'est question que de cela.

vous le savez, c'est un vrai sujet, dans la Sarthe comme ailleurs. Ce PLFSS ne répond malheureusement pas à la détresse de nos concitoyens. Je vous avais déjà interpellée l'été dernier quant au problème de l'accès aux soins, notamment à l'IVG, qui a déclenché une vive polémique médiatique.

Face à la désertification médicale, aux délais de rendez-vous de plus en plus longs et à la pénurie de spécialistes, la majorité promet des mesures incitatives. Pourtant, comme le démontre le rapport de la commission d'enquête sur l'égal accès aux soins, aucune des multiples mesures incitatives des dernières décennies n'a fonctionné. Nos collègues députés ont déjà proposé cet amendement, en vertu duquel, dans les zones présentant un fort excédent en matière d'offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s'installer en étant conventionné à l'assurance maladie que lorsqu'un médecin libéral de la même zone cesse son activité. leur avez répondu : « Le conventionnement sélectif n'a fonctionné nulle part en Europe, ni en Allemagne ni aux Pays-Bas, non plus qu'au Canada, en dépit des sommes phénoménales qui y ont été consacrées.

mais pourrait être contre-productive : sans négociation avec les professionnels de santé concernés, sans leur assentiment, ce dispositif pourrait détourner de jeunes médecins de l'exercice libéral, voire de l'exercice de la médecine tout court.

pourraient être raisonnablement envisagées lorsque l'installation du praticien n'a pas permis de remédier à la désertification, en dépit des propositions d'installation qui lui ont été faites. Ces mesures doivent se fonder sur l'évaluation établie par le directeur général de chaque ARS. Les conséquences de cette évaluation, aujourd'hui sans effet contraignant, pourraient faire l'objet d'un décret en Conseil d'État définissant les cas et les conditions dans lesquels, après concertation avec la profession, on pourrait décider de ne pas rembourser, ou de ne rembourser que partiellement les prestations assurées par des praticiens qui auraient refusé jusqu'à trois propositions successives d'installation. à travers cet amendement, pour remédier aux inégalités d'accès aux soins. Il suffit de mettre fin au bricolage de mesures et de tenir un discours ferme et clair afin de respecter l'égalité des territoires. La dématérialisation des consultations ne peut être qu'une réponse d'appoint. Les ruraux ou les périurbains ne doivent pas servir de cobayes à la robotisation de la médecine. Le rapport de notre collègue député Philippe Vigier, déposé en juillet dernier, se prononce très clairement pour des solutions de régulation. Cette mesure est d'intérêt général, et le législateur que nous sommes se doit de proposer des réponses concrètes aux Français qui n'ont pas, ou qui n'ont plus, accès aux soins.

des besoins en médecins région par région, afin de travailler à une meilleure couverture médicale en France.

Cohen, sur l'article. Cet article vise à permettre aux maisons de santé pluriprofessionnelles constituées en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires de salarier des auxiliaires médicaux en pratique avancée, afin d'accompagner le développement de ce mode d'exercice.

une complémentarité entre l'exercice en ville, les hôpitaux, les centres de santé et les maisons de santé. Nous ne les opposons pas.

n° 12 rectifié. L'article 31 entend permettre le salariat d'auxiliaires médicaux par les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, structures juridiques des maisons de santé. Dans l'exposé des motifs du projet de loi, il est noté que les professionnels de santé souhaitent une diversification de leur mode de rémunération au sein des structures libérales. Cette interprétation est fausse, si l'on en croit toutes les enquêtes menées auprès des étudiants en santé et des professionnels eux-mêmes. L'exercice libéral en maison de santé est l'un des premiers arguments en faveur d'un choix d'installation.

Enfin, l'argument selon lequel le salariat d'auxiliaires médicaux par les SISA permettrait d'améliorer l'accès aux soins est une aberration. À ce jour, l'exercice salarié de l'ensemble des auxiliaires médicaux est dans une situation critique en raison de l'absence de revalorisation de leurs grilles salariales. Cet article prônant le salariat risque donc de provoquer

éminemment dépendantes du type de structures existant déjà sur le territoire où elles souhaitent vivre. Dans certains cas, elles trouveront des centres de santé ; dans d'autres, des maisons de santé pluriprofessionnelles où tout le monde exerce en libéral. Si elles veulent être salariée d'une équipe médicale, pourquoi pas ?

Les structures des maisons de santé pluriprofessionnelles ont vraiment été pensées pour promouvoir l'exercice libéral. Cet amendement tend à en changer complètement la philosophie,

à lever les doutes sur la responsabilité d'un pharmacien qui ne reporterait pas le numéro RPPS du médecin prescripteur ou l'identifiant de sa structure d'exercice

à M. Alain Houpert. La télémédecine va permettre de pallier la carence de professionnels de santé dans certains territoires. On ne peut que s'en réjouir. Néanmoins, il convient que l'exercice de cette médecine à distance soit précisément encadré, afin d'offrir aux patients une qualité de diagnostic. Cela concerne, notamment, la téléradiologie, instaurée par la loi HPST de Mme Bachelot. Flairant la bonne aubaine, des sociétés situées au diable vauvert sont apparues pour proposer des actes de téléradiologie, qui sont préoccupants à plusieurs niveaux. Les patients

ainsi que je l'avais expliqué devant vous il y a exactement un an. On doit déplorer que nos collègues de l'Assemblée nationale n'aient pas pris la mesure de cette nécessité.

d'un guide des bons usages et de la qualité des actes de télémédecine. Ses travaux devraient m'être rendus au début de l'année 2019 et comprendront une partie sur l'imagerie médicale. Les

Mme la ministre. Lors de la remise du rapport de M. Cédric Villani, le Président de la République s'est engagé à développer l'intelligence artificielle dans deux champs prioritaires : la médecine et les transports. Mon ministère a été chargé de proposer une organisation qui permette de centraliser toutes les données de santé. Nous construisons

une fois l'arrêt de travail électronique établi, le prescripteur doit imprimer la notice d'information et remettre les documents papier au patient.

? L'article 32 prévoit que les régimes de sécurité sociale ont l'obligation de mettre à la disposition des prescripteurs des services leur permettant de prescrire des arrêts de travail de manière

par le vieillissement de la population active lié au décalage de l'âge de départ à la retraite : il s'agit de l'augmentation du nombre d'arrêts de travail longs, souvent liés à des pathologies chroniques. Cette partie-là du phénomène, nous la considérons comme totalement légitime. Seulement, nous constatons aussi une augmentation des arrêts de travail de

d'améliorer la capacité de contrôle de ceux qui veulent contrôler un certain nombre d'arrêts de travail. Quand vous recevez au bout de trois jours des arrêts de travail qui en font quatre, vous n'avez plus le temps de diligenter un contrôle. Cette instantanéité de l'information est donc importante si l'on veut réduire un certain nombre de pratiques.

Ce document permet de voir les ratios d'indemnités journalières prescrites par médecin, en fonction de la population. Avec la modélisation, on arrive véritablement à

en dehors de l'activité professionnelle. La notion d'activité autorisée ou non autorisée pendant les arrêts de travail n'est pas juridiquement définie. Il peut s'agir d'activités de loisirs, d'activités sportives, politiques ou sociales, voire familiales. À ce propos, la Cour de cassation a interprété les dispositions du code de la sécurité sociale comme interdisant à un salarié en arrêt de travail pour une maladie ou un accident d'exercer toute activité qui n'aurait pas été expressément autorisée par son médecin, sous peine de devoir restituer les indemnités journalières perçues. Or, même si de nombreux médecins encouragent les personnes arrêtées à mener des activités extraprofessionnelles, rares sont ceux qui l'inscrivent noir sur blanc sur les arrêts de travail. L'indemnité journalière a pour objectif d'assurer des revenus au salarié qui ne peut plus travailler, parce qu'il est malade ou victime d'un accident. Dans ce contexte, il paraît logique qu'il ne puisse cumuler ses indemnités avec les revenus d'une activité professionnelle. Toutefois, rien ne justifie d'exclure la possibilité d'exercer toute autre activité, celle-ci pouvant même être bénéfique pour l'amélioration de la santé du salarié et accélérer sa reprise d'activité professionnelle. C'est le cas notamment pour les arrêts liés à une affection

je vous remercie

ou en énumérant certaines activités autorisées, il ne peut pas dresser la liste exhaustive des activités autorisées patient par patient : cela augmenterait considérablement sa charge administrative.

qui permet une prise en charge renforcée par l'assurance maladie obligatoire et complémentaire des frais optiques, aides auditives et prothèses dentaires. L'annonce de ce dispositif a suscité de grands espoirs, car ces trois postes de dépenses de santé sont très faiblement remboursés par la sécurité sociale. Ils induisent donc à eux seuls des phénomènes de renoncement aux soins- entre 10 % et 35 % de la population, selon

tarifaire. Cette ouverture n'étant possible que par le recours à des complémentaires santé, on peut raisonnablement craindre que cette hausse des coûts ne soit répercutée, soit l'augmentation des tarifs des contrats, soit la réduction des paniers de soins proposés. Cette crainte est d'ailleurs confirmée par les nombreuses études de cabinets de courtiers portant sur le dispositif : elles annoncent une hausse des coûts de 7 % à 10 %. Certes, les complémentaires se sont engagées à ne pas augmenter leurs prix, mais quels mécanismes permettront de contrôler le respect de leurs engagements ?

Je veux bien vous croire, mais, actuellement, il existe déjà des dispositifs visant à permettre aux personnes en situation de précarité d'accéder à une protection complémentaire. Pourtant, elles sont des millions à ne pas avoir recours à leur droit à cette protection, et rien n'indique que cette situation change.

à une problématique majeure : l'accès aujourd'hui insuffisant à trois types de prestations. Il suffit d'avoir à l'esprit les restes à charge après intervention des complémentaires : 22 % pour l'optique, 25 % pour les soins prothétiques dentaires, 56 % pour les aides pour les aides auditives. Le dispositif prévu devrait redistribuer un milliard d'euros à l'ensemble de nos concitoyens, dont les deux tiers pris en charge par l'assurance maladie. Toutefois, il est vrai que des questions

quel sera le comportement des patients ? Comment vont-ils juger de la qualité de ce panier de soins ? Toutes les personnes âgées qui devraient être équipées d'un matériel d'audioprothèses vont-elles se précipiter chez les audioprothésistes

Les complémentaires sont aujourd'hui plutôt rassurantes sur le sujet. Néanmoins, une question précise se pose : celle des personnes allocataires de ce qu'on appelle les petits contrats,

monsieur le président, car je vois le temps passer ! -porte sur le plancher, qui sera modifié, pour les contrats responsables, en particulier dans le domaine de l'optique. De façon paradoxale, des personnes qui bénéficient aujourd'hui d'équipements d'un certain niveau verront leur reste à charge augmenter

toujours ! -cohérente : vous choisissez de changer notre système de santé et de décroiser les complémentaires de l'assurance maladie. Nous avons décidé de proposer cette offre dans le cadre du système français, dans lequel l'assurance maladie rembourse environ 75 % des dépenses de santé et les complémentaires les 25 % restants. Nous nous sommes inscrits dans ce système et avons donc réparti

en quelque sorte « bénéficié » du fait que nous vivons plus longtemps, avec davantage de pathologies chroniques : de plus en plus de malades en ALD

ne voudraient pas le « 100 % santé » mais souhaiteraient accéder à une offre de lunettes libre- je parle des montures -verront leur plafond de remboursement diminuer de 50 euros. C'était une façon d'absorber le coût de la réforme : nous avons cherché des équilibres globaux,

le projet de nomenclature sur le « 100 % santé », en discussion entre votre ministère et les représentants des opticiens, prévoit la transmission au patient d'un questionnaire de satisfaction, qui lui sera adressé en dehors du magasin, une fois l'équipement correcteur acquis. L'opticien ne pourra ainsi pas participer à ce dispositif d'évaluation de la délivrance de l'offre « 100 % santé », tel qu'il est prévu à l'alinéa

rapporteur. Le projet de loi prévoit un dispositif de sanction en cas de non-respect par les fabricants ou les distributeurs des obligations instituées par le texte pour la mise en oeuvre des

et des règles en matière de présentation des devis. En effet, les contours du dispositif d'évaluation ne sont pas assez clairement définis pour permettre d'apprécier le rôle joué par les distributeurs dans sa mise en oeuvre. En outre, l'article L. 165-9-1 du code de la sécurité sociale fixe déjà une amende administrative en cas de manquement aux obligations relatives à la présentation des devis. Quel est l'avis du Gouvernement

devis. Sinon, les Français n'y accéderont pas et ce droit ne sera que formel. Si nous supprimons toute sanction, nous pouvons être quasiment certains que les devis ne comprendront pas d'offre « 100 % santé L'objectif est non pas de sanctionner, mais de mettre en oeuvre une nouvelle façon de pratiquer l'accès à l'offre de soins en prothèses auditives ou en lunettes.

Le texte du projet de loi ouvre la possibilité de déroger à la procédure « classique » de négociation des tarifs de responsabilité des produits et prestations éligibles au remboursement par l'assurance maladie, fixés par convention entre le fabricant ou le distributeur de santé, ou, à défaut, par décision de ce comité. Par dérogation, les tarifs des produits hors panier « 100 % santé » pourraient être fixés par arrêté ministériel. Nous avons souhaité supprimer la possibilité de fixation unilatérale des tarifs, car la commission préfère privilégier, d'une manière générale, les procédures de conventionnement entre les

Mais, dans le cas présent, il nous semble qu'une procédure simplifiée par arrêté est pleinement justifiée. Dans le secteur de l'optique, les bases de remboursement par par la sécurité sociale des équipements hors « 100 % santé » seront tellement faibles et symboliques qu'il est préférable de passer par un forfait. Cela ne mérite pas une négociation conventionnelle entre les lunettiers et le CEPS. Nous pensons qu'il n'y a pas d'enjeu de négociation vu des sommes en jeu. Nous préférons donc que les tarifs soient fixés forfaitairement par les ministres. Mais je peux vous rassurer, la voie conventionnelle reste bien la voie de droit commun pour tous les dispositifs médicaux. Dans le cas précis de l'optique, en dehors du « 100 % santé », elle n'a pas de justification. Je vous demande donc de retirer votre amendement ; à défaut, j'y serai défavorable.

M. Philippe Mouiller. Par cet amendement, il est proposé que tout devis remis par un professionnel de santé à un assuré lors de la vente comporte obligatoirement les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance maladie complémentaire. Dans le cadre de la mise en place du « 100 % santé », ces organismes complémentaires se sont engagés à améliorer la lisibilité des contrats et leur comparaison, afin de faciliter un choix éclairé du consommateur. éclairé du consommateur. Ainsi, tous les contrats comporteront un tableau de garanties avec des libellés communs pour les grands postes de soins et un tableau d'exemples de remboursement en euros. Toutefois, l'absence de caractère contraignant de la mesure limite l'impact de cet engagement.

dans cet article améliore la lisibilité des contrats, puisque, en l'état, l'obligation reposerait sur les professionnels assurant la distribution des produits et non sur les complémentaires. Je demande donc le retrait de cet amendement

sous la forme de nouvelles décisions unilatérales des employeurs ou d'accords collectifs d'entreprise renégociés, afin de pouvoir continuer à bénéficier des exonérations sociales liées aux contrats de frais de santé. En effet, si les entreprises ne respectent pas l'échéance du 1 janvier 2020, elles perdent, d'une part, le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations du financement patronal, et, d'autre part, l'application du taux réduit de taxe de solidarité additionnelle, la TSA, fixé à 13,27 %, ainsi que le crédit d'impôt de TSA dans le cadre de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé.

Certains appellent à une appréciation bienveillante pour l'année 2020. Il est par ailleurs nécessaire que les décrets paraissent tôt, pour laisser le temps de faire les adaptations nécessaires. Il est vrai que le report d'un an, tel que proposé, conduirait à différer d'autant l'entrée en vigueur de la réforme. Nous souhaiterions connaître l'avis du Gouvernement, pour obtenir des assurances quant à ces modalités d'entrée en vigueur. Quel est Les décrets seront publiés à la fin de l'année 2018. L'amendement que vous proposez, monsieur Morisset, n'est conforme ni à la négociation que j'ai menée avec l'ensemble des parties prenantes ni aux engagements que j'ai pris devant les Français. Je ne peux y être que défavorable.

aura pour objectif d'évaluer la mise en oeuvre de la réforme et ses effets, tant sur les marchés concernés que sur le recours aux soins ou encore sur les niveaux de couverture complémentaire. Il réunira la totalité des acteurs concernés par la réforme : les représentants des organismes complémentaires de l'assurance maladie, les assurés, les fabricants et les distributeurs. Il est prévu dans le décret que le comité nous remette un rapport tous les deux ans, portant notamment sur les pratiques constatées et dressant un bilan de la mise en oeuvre des réformes. Je sais votre Haute Assemblée soucieuse d'éviter les rapports inutiles. Votre proposition étant satisfaite, nous vous suggérons de retirer votre

Guyane. Des financements sont octroyés chaque fin d'année dans certains établissements, en raison des difficultés de trésorerie. Il serait important pour nous de prendre en compte ces difficultés

Le fait de préciser dans la loi les principaux facteurs à prendre en compte pour la définition des coefficients de majoration des tarifs outre-mer ne sera pas forcément la garantie d'une réponse efficace aux problèmes réels qui se posent. Néanmoins, il est vrai qu'une évaluation précise des besoins et de la situation dans chaque territoire serait nécessaire. Partageant cette préoccupation, la commission a émis un avis de sagesse. Quel est

penser l'équilibre du budget des hôpitaux des DOM n'est pas la bonne formule. D'abord, parce que chaque hôpital et chaque département souffrent de problématiques diverses par exemple, à la Martinique, nous savons que la déprivation démographique est un facteur important de diminution de l'activité. On pourrait toujours augmenter les tarifs, mais il faudrait, en réalité, redimensionner l'hôpital, y compris en termes de structures, pour s'adapter à une population quelque peu différente de ce qu'elle était au moment où l'hôpital a été construit. De la même façon, certains établissements font face à des difficultés de prise en charge de populations très particulières, qui sont mal identifiées par la tarification à l'activité, la T2A. Or le coefficient géographique ne s'applique les GHS, et à la T2A. Nous pensons, au contraire, qu'il faut diversifier les modes de rémunération de ces établissements, pour qu'ils puissent prendre en charge correctement un certain nombre de pathologies spécifiques. Je pense notamment à Saint-Martin, qui connaît des problématiques très importantes d'addictions, de grossesses précoces, etc. Aujourd'hui, nous sommes très attentifs aux questions de tarification dans les DOM. J'ai d'ailleurs demandé à la mission de Jean-Marc Aubert, qui travaille sur les nouveaux modes de tarification des hôpitaux, d'inclure une réflexion spécifique sur les DOM